La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 4 décembre 2024 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n’y a pas d’observation

Messieurs les ministres, mes chers collègues, le cyclone Chido a durement frappé, en le traversant de part en part, le département de Mayotte, laissant derrière lui un paysage de désolation. À des dégâts considérables s’ajoute un bilan humain dont nous ne connaissons pas encore l’ampleur, en nombre de blessés et de pertes humaines, en raison de l’étendue de de l’habitat informel et des grandes difficultés d’accès. Compatissant à la douleur de nos compatriotes mahorais, je tiens à leur exprimer au nom du Sénat tout entier notre solidarité et notre soutien, à les assurer de notre mobilisation à leurs côtés pour les aider à surmonter cette terrible épreuve. J’assure toutes les familles, en particulier celles qui ont perdu un proche et dont le courage et la résilience forcent le respect, de notre profonde sympathie. J’ai une pensée particulière pour nos collègues sénateurs de Mayotte, Salama Ramia et Saïd Omar Oili, avec lesquels je

le préfet, le président du conseil départemental, les forces de secours et de sécurité et les acteurs de la sécurité civile et de la santé, ainsi que les militaires, tous mobilisés pour venir en aide à la population dans des conditions extrêmement difficiles. L’heure est à l’urgence pour permettre à nos compatriotes, si attachés à la République, en particulier aux nombreux enfants isolés, de disposer d’eau, de nourriture, d’un toit pour s’abriter et de l’accès aux soins. Les communes, sur lesquelles s’appuie l’État, jouent un rôle essentiel dans ce dispositif. Je salue l’engagement des maires et de l’ensemble des élus, qui, comme toujours lors des crises, sont en première ligne pour apporter un soutien immédiat à la population et pour aider leurs collectivités à surmonter cette épreuve. Lorsque viendra le temps de la reconstruction, nous devrons réfléchir avec les élus locaux à une solution durable tenant compte de la situation des Mahoraises et des Mahorais, du département et de son environnement régional.

Mes chers collègues, c’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès soudain de notre ancien collègue Roger Madec, qui fut sénateur de Paris.

Il fut également vice président du conseil régional d’Île de France. Élu sénateur en septembre 2004, puis réélu en septembre 2011, il siégea naturellement au sein du groupe socialiste.

Au sein de notre institution, il travaillait notamment sur les questions relatives aux droits des collectivités territoriales. Nous nous souvenons de son investissement lors des débats de société qui marquèrent son mandat, notamment ceux sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe.

qui fit beaucoup pour son arrondissement. Je veux assurer sa famille et ses proches de notre sympathie et leur présenter nos condoléances les plus sincères.

recueillement. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie le mercredi 11 décembre 2024, sont consultables sur le site du Sénat.

l’arrivée de notre nouveau collègue, Jean Marc Ruel, sénateur de Saint Pierre et Miquelon. Au nom du Sénat tout entier, je lui souhaite la bienvenue dans notre assemblée. L’ordre L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi spéciale

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous n’ignorez pas qu’une motion de censure, adoptée le 4 décembre dernier lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, a interrompu la discussion des textes financiers, qu’elle a compromis l’adoption d’une loi de finances pour 2025 et qu’elle a, pour le moment, privé notre nation d’un budget. J’ai eu l’occasion de le dire en commission des finances, et je le répète ici, cette situation est grave et exceptionnelle.

conformément à l’engagement pris par le Président de la République devant les Français le 5 décembre dernier. Il n’est donc – je le répète – qu’un texte technique, sans portée politique, qui vise uniquement à éviter la discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption

dans une limite maximale, qui est celle du budget de l’année précédente. En aucun cas nous ne pouvons dire – donc nous en satisfaire – que cette loi permettrait de passer une année.

: premièrement, continuer à lever l’impôt, permettre de tenir nos engagements, notamment à l’égard de l’Union européenne, et donner de la visibilité aux collectivités locales ; deuxièmement, permettre à l’État et aux organismes de sécurité sociale de continuer à émettre de la dette. Aujourd’hui, notre responsabilité collective est donc contenue contenue à l’examen et à l’adoption de cette loi spéciale que nous vous soumettons. Je veux saluer ici, bien sûr, l’esprit de responsabilité dont a fait preuve l’Assemblée nationale en adoptant ce texte à l’unanimité des 481 députés votants. Je ne doute pas que le Sénat fera de même.

Le projet de loi spéciale que vous vous apprêtez à examiner ne saurait en tenir lieu. Le Premier ministre l’a lui même clairement souligné, lors de la passation de pouvoir vendredi dernier et, de nouveau, hier lors de la séance de questions La situation de nos finances publiques n’a pas changé depuis la censure du Gouvernement. L’état de nos comptes est le même, avec tous les défis que cela emporte pour le présent comme pour l’avenir. La décision de l’agence de notation Moody’s, ne nous dit pas, hélas ! autre chose. Chacune et chacun ici – je le sais – en est parfaitement conscient. Malgré l’issue des débats budgétaires, il ne s’est trouvé personne, sur quelque travée que ce soit, pour contester la gravité de la situation, le caractère excessif de notre endettement ou la nécessité de réduire le déficit. Il y a donc au Parlement, je le crois, un espace pour engager le redressement des comptes publics, pourvu que les forces politiques qui le composent parviennent à s’entendre, en responsabilité, sur les modalités de l’effort à fournir. Ce texte ne préjuge donc pas des nouveaux arbitrages qui seront rendus, sous l’autorité de François Bayrou, par un prochain gouvernement de plein exercice. Il ne préempte en aucun cas les futures décisions budgétaires, dont je souhaite évidemment qu’elles soient prises rapidement, dans l’intérêt supérieur de notre pays et de nos concitoyens.

En premier lieu, la loi spéciale ne permet pas de modifier le code général des impôts. Elle n’exprime pas le consentement à l’impôt ; elle n’en constate que la nécessité. Elle ne permet donc ni de reconduire pour l’année suivante les dispositions fiscales qui arrivent à échéance à la fin de l’année 2024

Cette loi spéciale ne peut qu’autoriser temporairement le Gouvernement à continuer à percevoir les impôts et taxes existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. C’est indispensable pour assurer le financement de nos services publics, de notre système de protection sociale et, bien sûr, des collectivités territoriales. En second lieu, le décret qui sera pris après la promulgation de la loi spéciale nous place sous le régime restrictif des services votés. La loi spéciale n’autorise pas le Gouvernement à engager des dépenses nouvelles. Conformément à la Constitution et jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi de finances pour l’année, les crédits se rapportant aux services votés seront donc temporairement ouverts par décret. Ces services votés correspondent au niveau minimal de crédits jugé indispensable pour permettre l’exécution des services publics en 2025 dans les conditions de l’année précédente.

Sauf nécessité pour la continuité de la vie nationale ou motif d’urgence caractérisé, le Gouvernement ne pourra pas non plus procéder à de nouveaux investissements ou à des dépenses discrétionnaires de soutien aux associations, aux entreprises ou aux collectivités.

Enfin, la loi spéciale autorise le Gouvernement à recourir aux emprunts nécessaires pour assurer ses engagements, ainsi que le fonctionnement régulier des services publics. Vous le savez, les recettes fiscales et sociales ne suffiraient pas à couvrir le besoin de financement des administrations publiques ; c’était d’ailleurs tout l’objet des débats sur la dette Nous ne pourrions donc pas assurer nos engagements auprès de nos créanciers ni garantir le fonctionnement régulier des services publics sans la possibilité de recourir à l’emprunt. Par conséquent, il est indispensable d’autoriser tant l’État que les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et l’Agence centrale des

Il s’agit d’assurer la continuité de la Nation, le fonctionnement régulier des services publics et le respect des engagements pris par notre pays. Avec ce texte, nous vous proposons tout simplement que nécessité fasse loi, dans le respect du droit. La parole

Sous la V République, en effet, jamais la France n’a connu une telle situation budgétaire. La toute récente censure politique nous a rendus incapables de nous doter d’un budget pour l’année à venir ; nul ne sait à cet instant quand nous serons en mesure d’en voter un.

Nous ne sommes pas réunis aujourd’hui pour en déterminer les responsabilités, mais il me semble que notre pays n’avait pas besoin de cela, et nos finances publiques encore moins. La vérité, c’est que la France se retrouve dans une situation de très grande fragilité.

celle ci reste relativement élevée, et l’on peut trouver plusieurs raisons de se rassurer en constatant que le avec l’Allemagne n’augmente pas davantage ou que le CAC 40 continue de progresser. Mais ne nous voilons pas la face l’incapacité de la France à se doter d’un budget est très grave, même si elle n’a pas à court terme les conséquences catastrophiques que certains veulent lui donner. Les deux précédents que nous avons connus sous la V République n’ont rien à voir avec la situation actuelle, puisque, tant en 1962 qu’en 1979, le Parlement avait très vite voté un budget au début de l’année suivante. La France ne faisait alors pas face à l’instabilité politique. Comment savoir

Par ailleurs, le taux de chômage repart à la hausse et reste sensiblement supérieur à celui de la zone euro, alors que le nombre de défaillances d’entreprises est au plus haut. Enfin, le déficit commercial de la France demeure lui aussi abyssal, à plus de 80 milliards d’euros sur les douze derniers mois, tandis que notre dette publique tutoie des sommets vertigineux. Compte tenu du contexte inédit et très dégradé dans lequel nous avons à examiner ce projet de loi spéciale,

une censure gouvernementale empêchant la promulgation d’une loi de finances avant la fin de l’année, ne correspond pas strictement aux procédures d’urgence prévues dans ces textes. Malgré la qualité de notre cadre constitutionnel et organique, nous sommes dans un cas de figure qui n’a pas été prévu par les textes. J’y reviens, il est grave de se trouver dans une telle situation institutionnelle.

dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures d’ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale. » Cette jurisprudence est confirmée par l’avis du Conseil d’État rendu récemment à la demande du Gouvernement.

La vie nationale doit continuer, mais toutes les mesures qui ne seraient pas strictement « nécessaires » à cette poursuite n’ont pas leur place dans ce texte. À cet égard, je vous avoue que le débat sur l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu m’a rendu perplexe. Cette indexation n’est évidemment pas nécessaire à la continuité de la vie nationale. Pour autant, elle se fera, et le Gouvernement nous a confirmé que nous disposions de plusieurs mois pour la voter. Je vous propose donc de sortir ce sujet du projet de loi spéciale qui nous occupe.

Cela permettrait de nous donner à la fois un cap et une boussole pour 2025, en entamant le redressement de nos comptes qui est si nécessaire. Indexation du barème de l’impôt sur le revenu, mesures pour les agriculteurs, trajectoire de la loi de programmation militaire, etc. Je souhaite que, face aux enjeux auxquels notre pays doit faire face, un sursaut nous permette d’unir nos forces rapidement pour parer ces risques immédiats et agir face à l’urgence.

Parce que ces articles paraissent nécessaires et suffisants et parce que la priorité est de rassurer les Français en garantissant la poursuite de la vie nationale, la commission des finances propose d’adopter ces quatre articles sans modification,

Il s’agira d’un enjeu essentiel durant les semaines à venir. Ces crédits correspondent au minimum indispensable pour poursuivre l’exécution des services publics. Avant la Lolf, le montant des services votés figurait dans le projet de loi de finances ; ce n’est plus le cas aujourd’hui.

les services votés seront ouverts sans autorisation parlementaire, puisque nous n’avons pas voté de loi de finances initiale. Toutes ces raisons doivent nous pousser à poursuivre et à achever rapidement l’examen du projet de loi de finances pour 2025 en cours de discussion.

avec force, cette loi spéciale donnera tout ce qu’il faut à l’État pour assurer ses fonctions essentielles au début de 2025, mais rien de plus. plus. Il nous faut le plus rapidement possible achever l’examen du projet de loi de finances en cours de discussion, afin de donner un budget à notre pays et de rassurer les Français. Enfin, notre responsabilité est aujourd’hui de nous unir, en mettant de côté nos divergences et en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur de notre pays et des Français. Cet intérêt supérieur, nous le servirons ensemble, en rassemblant nos forces, pour participer au redressement de nos comptes publics et retrouver la confiance en l’avenir. La parole

Nous voilà donc réunis, en ce début d’après midi, pour examiner un nouveau type de loi : la loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique relative

La loi spéciale a, comme vous le savez, le statut de loi de finances. La commission des affaires sociales s’est saisie pour avis de l’article 3, qui autorise la sécurité sociale à emprunter.

La disposition des lois de financement de la sécurité sociale autorisant la sécurité sociale à emprunter comprend des plafonds pour les différents organismes concernés. Par exemple, dans le cas du PLFSS pour

Lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur un amendement du rapporteur général tendant à rétablir ces plafonds. Le ministre chargé du budget et des comptes publics a justifié cet avis en arguant que, selon lui, de tels plafonds politiques n’auraient pas relevé du champ de la loi spéciale et n’auraient donc pas été constitutionnels. Que l’on partage ou non cette analyse, il serait paradoxal d’introduire des plafonds d’emprunt, par nature politiques, dans un texte censé être purement technique. Cette absence de plafonds s’explique aussi probablement par des raisons pratiques.

il avait fallu mettre en place un financement d’urgence impliquant la Caisse des dépôts. Comme la Cour des comptes l’a récemment rappelé, le financement des déficits par l’Acoss se fait « dans des conditions qui pourraient mettre en risque le versement des prestations ».

ce qui n’aura de sens et ne sera possible que si on sait où l’on va et donc si l’on dispose d’une loi de financement de la sécurité sociale, avec une programmation crédible.

indispensable pour assurer le financement nécessaire au fonctionnement des institutions et des services publics. Je me réjouis que l’Assemblée nationale l’ait adoptée à l’unanimité, ce que s’apprête probablement à faire le Sénat si les votes constatés en commission des finances se confirment.

Cela conduit à ce que ne soient permises que des mesures d’ordre financier « nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale », comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel.

Aussi, face aux choix qui s’offrent à nous, j’estime, comme le rapporteur général, que la poursuite de la discussion du projet de loi de finances que nous étions en train d’examiner constitue la meilleure solution, parce que c’est la plus rapide et la plus efficace. Évidemment, la copie initiale du gouvernement démissionnaire doit être revue pour mieux traduire les aspirations profondes des Français, qui se sont notamment manifestées lors des dernières élections législatives. Toutefois, la procédure parlementaire permet

finir l’examen du texte en première lecture, puis l’Assemblée nationale en débattre dans le cadre d’une deuxième ou d’une nouvelle lecture. Durant ce travail parlementaire, rien n’empêchera le gouvernement nouvellement installé de proposer lui même des modifications, y compris

plutôt que de nous embarquer dans l’élaboration d’un nouveau texte, qui, en raison de la préparation technique et du travail parlementaire qu’elle impose, exigerait un délai de plusieurs mois, nous devons choisir, ensemble, le pragmatisme et l’efficacité.

et même dommageable pour notre pays –, il nous resterait toujours la possibilité d’adopter, au travers d’un texte législatif autonome, les mesures fiscales les plus attendues par nos concitoyens et apportant les correctifs les plus importants. Une proposition de loi indexation du barème de l’impôt sur le revenu est déjà prête et pourrait être rapidement déposée par le rapporteur général et moi même ; d’autres mesures pourraient éventuellement y être associées.

En effet, si nous examinons ce texte aujourd’hui, c’est précisément parce que le précédent gouvernement, auquel vous apparteniez, messieurs les ministres, a refusé de voir les réalités politiques du pays. Depuis deux ans, Emmanuel Macron se comporte comme un mauvais perdant, qui veut sans cesse rejouer le match qu’il a pourtant perdu, et par trois fois ! Il sera le président qui n’aura jamais été capable de tirer les leçons de ses défaites : tel un joueur de poker compulsif,

Dans quelle démocratie saine le Premier ministre est il issu de l’un des plus petits groupes de l’Assemblée nationale ? Dans quelle démocratie saine le Président de la République utilise t il son pouvoir de nomination comme un pouvoir de décision, faisant fi de tous les enseignements des différents scrutins ? Ce piétinement des résultats n’est pas sans conséquence pour le pays. Les études sur le sujet mettent en relief des chiffres désastreux, qui témoignent à eux seuls du climat de défiance qui règne dans le pays. En deux décennies de règne, après huit guerres de religion, Henri IV changea de religion à six reprises et réconcilia entre eux les Français, tout en redressant le pays. Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, qui se voit volontiers comme un Henri IV moderne, a la lourde tâche de réconcilier entre

ne changera rien… Pour réussir à réconcilier le pays, il va falloir l’écouter et entendre ce qu’il nous a dit lorsque le Président de la République a mis en œuvre sa « dissolution d’amertume » en juin dernier. Quel est l’intérêt de redonner la parole au peuple si c’est pour ne tirer aucune conséquence politique quand ce dernier s’est massivement exprimé ? Il est clair que, par cette nomination, le Président de la République préfère la coalition à la cohabitation. À tous ceux qui nous disent que la personnalité du nouveau Premier ministre, conjuguée aux conditions pour le moins baroques de sa nomination, garantira une cohabitation, je tiens à rappeler un principe simple : la cohabitation, c’est lorsque le parti du Président de la République est dans l’opposition. Tout le reste n’est que littérature… En dépit de ce nouveau coup de force d’un macronisme finissant, le gouvernement sur le point d’être nommé sera presque celui de la dernière chance pour Emmanuel Macron. Le président qui se voyait en maître des horloges devrait entendre le compte à rebours qui est désormais lancé, car, au delà des dégâts inhérents de la politique promue par Emmanuel Macron, ce qui est désormais en cause, ce sont les dégâts que sa conduite entraîne. Nous arrivons à un moment où sa manière d’exercer le pouvoir représente un coût astronomique pour les Français.

Je le dis donc avec gravité et solennité, le prochain gouvernement devra changer de méthode de travail par rapport au gouvernement censuré, sans quoi les mêmes causes produiront les mêmes effets. À ce titre, je tiens à dire publiquement que le groupe socialiste n’a pas goûté la salve d’amendements visant à supprimer plusieurs mesures emblématiques adoptées par la Haute Assemblée durant l’examen du budget. En moins de deux heures, vous avez, messieurs les ministres, rayé d’un trait de plume des mesures pourtant adoptées par le Sénat, telles que la hausse de la, de l’ ou de la taxe dite

Le changement de méthode doit donc avoir lieu, et très vite, car sept ans de macronisme ont mis les finances publiques dans un état de délabrement qui ne nous permet plus d’attendre.

il semble désormais capital de mettre un terme à l’instabilité politique qu’a lui même créée le président Macron, tout en gardant la mesure nécessaire qui incombe aux fonctions respectives des uns et des autres. Les tentatives de dramatisation, frôlant parfois la malhonnêteté intellectuelle, n’ont pas eu prise sur un pays ayant besoin de sérénité. Je le rappelle, les marchés, tout comme nos concitoyens, veulent de la stabilité. Ils ne cherchent pas un champion de saut en hauteur…

Lors de son allocution télévisée, le chef de l’État a indiqué qu’il ne croyait pas que l’avenir de la France puisse se faire avec plus d’impôts. c’est bien avec moins de réductions des dépenses et plus de recettes fiscales que nous entendons engager le rétablissement de nos comptes publics. Les baisses d’impôts successives des sept dernières années nous ont coûté 62 milliards d’euros par an. Pilier fondamental du macronisme économique, le principe de ces suppressions de prélèvements obligatoires a donné les résultats que l’on sait : des dérapages budgétaires, une économie en panne de productivité, une compétitivité en berne. Pour bâtir un consensus parlementaire, les soutiens du Président doivent s’affranchir des dogmes du patron : la France se porte plus mal depuis les baisses d’impôts massives ; il vous faudra tôt ou tard le reconnaître, mes chers collègues, mon propos est résolument tourné vers les échéances budgétaires à venir, tant ce projet de loi spéciale n’appelle aucune réflexion particulière. En effet, ce texte de loi tampon se contente d’autoriser le Gouvernement à continuer de percevoir les impôts existants et à reconduire les dépenses de l’État au niveau de celles de 2024. Le groupe socialiste regrette vivement que l’amendement visant à indexer sur l’inflation le barème de l’impôt sur le revenu pour les tranches les plus basses ne satisfasse pas les règles de recevabilité financière.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, on retiendra que la dernière chose que sait faire l’État quand tout va mal, c’est de percevoir l’impôt avec précision et efficacité, quitte à rendre imposables 380 000 foyers supplémentaires. C’est une allégorie qui en dit long sur l’état de l’État ! La faute à qui ? Qui a censuré Les décisionnaires qui gouvernent et les fonctionnaires qui administrent auront réussi à étouffer tout dynamisme à l’intérieur du pays, tout en dispensant les bienfaits de l’État providence au monde entier, sans vouloir se rendre compte qu’ils pompaient un marais déjà asséché. Résultat, de déficits en dettes et de dettes en déficits, nous parvenons, après soixante six ans de V République et cinquante ans de budgets déficitaires, à une situation inédite : le blocage politique sur notre budget national en fin d’année civile. Ne prenez pas ce projet de loi spéciale pour un texte banal ou une formalité de gestion ; c’est un terrible avertissement. Le niveau de ras le bol des Français augmente aussi vite que leur niveau de vie diminue et aussi systématiquement que vous refusez de remettre en cause les dogmes ruineux des dernières décennies : toujours plus pour la Commission européenne, toujours plus pour l’assistanat, toujours plus pour l’immigration, toujours plus pour les administrations d’État… En 2019, les « gilets jaunes » avaient demandé simplement deux choses : qu’on leur donne la parole et qu’on leur permette de vivre dignement de leur travail. Au lieu d’un renouveau démocratique, vous leur avez imposé vingt cinq 49.3, un « front antirépublicain », des combines contre nature pour empêcher que le Gouvernement ne soit renversé et aucune évolution du référendum d’initiative partagée. Pour ce qui est de la juste rémunération du travail, vous n’avez su proposer qu’inflation, impositions et cotisations supplémentaires, pour pallier le « n’importe quoi qu’il en coûte ». Aucune remise en question, et une véritable autoroute de l’injustice qui mène nécessairement à un avenir bien sombre. Alors que Mayotte est entièrement détruite et que l’argent et les moyens manquent, vous confirmez cette provocation qui consiste à accorder, dans le cadre de l’aide publique au développement, 120 millions d’euros à la Chine, 171 millions d’euros à la Turquie et 800 millions d’euros à l’Algérie

le projet de loi spéciale que nous examinons cet après midi est le texte de tous les paradoxes ; vous en avez cité un, madame la rapporteure

alors que cette crise jette le discrédit sur l’ensemble de la classe politique, il est un roc qui résiste, ce sont nos institutions. Nous pouvons, cet après midi, adopter un texte permettant d’assurer la continuité de l’État, temporairement,

Cette Constitution et nos lois organiques, il nous appartient de les protéger ; c’est notre trésor, mes chers collègues. Très bien ! Alors même que certains, à l’Assemblée nationale, ont essayé de les contourner, notre bicamérisme

tout en protégeant notre trésor commun. C’est la démonstration que, dans les pires moments de notre histoire, les institutions de la V République fonctionnent et opposent des garde fous aux apprentis sorciers.

Gardons nous donc de nous amuser avec notre Constitution… Citons également Benjamin Constant, pour qui une Constitution est un pacte entre les générations et un rempart contre les passions du moment. Laissons donc, mes chers collègues, les passions du moment et concentrons nous sur l’intérêt général de la Nation et des Français.

devra être corrigé dans ces deux directions. Il devra également préserver l’investissement dans la défense, dans la justice, dans la sécurité, dans la santé et dans l’éducation. Alors que la société devient chaque jour plus violente et que la guerre fait tomber toujours plus d’obus sur l’Europe,

Monsieur le président, permettez moi d’associer l’ensemble des sénateurs du groupe Les Républicains à vos propos relatifs au département de Mayotte. Messieurs les ministres, mes chers collègues, le contexte politique de ces derniers mois a donné au Sénat un rôle de premier rang dans le cadre du débat budgétaire. Rarement, voire jamais, nos travaux sur un projet de loi de finances n’avaient été aussi suivis et considérés. Exercice constitutif de la souveraineté, le fait de lever l’impôt et d’en déterminer l’usage en dépenses est un principe constitutionnel mentionné à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce principe se matérialise dans la procédure budgétaire française, qui tend à confier au seul Parlement le vote du budget et la compétence fiscale. Toutefois, la rationalisation du pouvoir législatif entamée dès 1958, puis le virage de la Lolf à l’aube des années 2000, ont réduit la participation du Parlement en matière financière.

La discussion budgétaire en est naturellement amoindrie et se concentre trop souvent, malheureusement, sur la défense politique d’intérêts spécifiques, au lieu d’être consacrée aux enjeux globaux des finances publiques, à la pluriannualité ou à la responsabilisation.

Le contexte politique actuel offre au Parlement l’occasion de se saisir plus intelligemment de la question budgétaire, dans une logique de responsabilisation des pouvoirs publics. Le Gouvernement, mes chers collègues, a besoin de notre expertise, de notre appui et de notre soutien pour garantir l’adoption d’un budget sérieux et partagé. Ce nouveau cycle de travail commun commence aujourd’hui avec l’examen de ce projet de loi spéciale. Cette loi répond là encore à des exigences constitutionnelles. Je pense à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. S’y ajoutent les principes constitutionnels de continuité et d’égalité du service public. Voter cette loi est incontournable. Rejeter le texte serait irresponsable, pour les Français, mais aussi pour la France. Notre pays a besoin d’un cadre économique, budgétaire et financier. La France a besoin d’un budget.

Depuis la dissolution, notre écart de taux avec l’Allemagne s’est accentué. Si les marchés financiers ont peu réagi au vote de la motion de censure, c’est parce qu’ils avaient déjà fortement sanctionné la décision du Président

pour le service public et pour l’investissement ». Comment, à l’avenir, pourrons nous financer la transition écologique et rester compétitifs dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la santé si 100 milliards d’euros sont captés par le paiement des intérêts ?

2026. Il est grand temps d’être responsables. Nous devons rassurer les Français et les milieux économiques en adoptant rapidement un PLF au début de l’an prochain.

a été intégralement adoptée le 23 février de cette année là, ainsi que l’annulation de la loi de finances pour 1980 un jour de réveillon de Noël. Ces deux souvenirs pourraient nous laisser penser que la situation dans laquelle nous sommes ne serait en rien nouvelle. Pourtant, mes chers collègues, le moment est bel est bel et bien inédit, et cela pour trois raisons. Tout d’abord, il l’est compte tenu du contexte politique. Malgré la nomination d’un nouveau Premier ministre, le Gouvernement qui présente le présent projet de loi est démissionnaire, car il a été censuré par une majorité de 331 députés. L’hémicycle de l’Assemblée nationale est fragmenté, aucune majorité solide n’y existe à ce stade et sa dissolution est impossible dans l’immédiat. Ensuite, le moment est inédit, parce que les finances publiques placent la France dans une position difficile, où l’immobilisme serait fatal. car notre pays est doté depuis 2001 d’une loi organique qui encadre l’adoption de ce projet de loi spéciale. Mes chers collègues, je n’ai nul besoin de vous convaincre. Mais posons nous la question pour celles et pour ceux qui nous écouteraient depuis l’extérieur de notre assemblée pourquoi l’adoption d’un projet de loi spéciale est elle nécessaire pour le pays ? Un budget permet, en schématisant, l’autorisation de percevoir des recettes et de réaliser des dépenses. Or qui dit absence de budget dit aussi absence de recettes et de dépenses. Si aucun PLF n’est voté pour l’année à venir, en l’occurrence 2025, de quel droit l’État pourrait il continuer à percevoir les impôts ? Telle est la principale raison d’être de ce projet de loi spéciale : répondre à cette question par un texte transitoire, au contenu au contenu limité, mais vital pour notre pays et pour la continuité de nos services publics. Je précise bien : « au contenu limité », car le domaine de ce texte est strictement encadré, raison pour laquelle il ne contient que quatre articles. L’article 1 autorise l’État à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la prochaine loi de finances, sans en ajouter ni en retirer. L’objectif est de permettre à l’État, ainsi qu’aux autres personnes publiques, de percevoir de manière temporaire les ressources nécessaires pour assurer la continuité de leurs missions. Il s’agit également de rendre possible la reconduction des prélèvements sur les recettes de 2024 au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales, avec, pour ces dernières, le détail introduit par nos collègues députés à l’article 1 . Les articles 2 et 3 du projet de loi visent quant à eux à autoriser l’État à recourir à l’emprunt et à habiliter à habiliter les régimes et organismes de sécurité sociale à recourir à des recettes non permanentes, avec, en ligne de mire, la nécessité de couvrir leurs besoins de trésorerie. Je répète : « au contenu limité », du fait de la tentation d’introduire par voie d’amendement l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu.

est nécessaire pour nos concitoyens. Mais comme le Conseil d’État l’explique, notre droit, en l’occurrence la Constitution et la Lolf, ne permet pas d’intégrer cette mesure dans le projet de loi spéciale. L’indexation doit être décidée par notre Parlement dans le cadre de la future discussion budgétaire et fiscale, car il s’agit d’une décision

regrettables pour les embauches. Elles se font sentir également pour nos concitoyens de Nouvelle Calédonie, qui devront attendre le milliard d’euros annoncé face aux dégâts causés par les émeutes. Elles pèsent sur nos agriculteurs, qui patienteront encore pour les nombreuses mesures de soutien fiscal dont ils auraient pu bénéficier bien plus tôt. pas non plus que cette censure a accéléré la première étape de conclusion des négociations du traité de libre échange entre l’Union européenne et le Mercosur, un traité auquel s’opposent largement le Parlement et,, le pays.

de dégrader la note souveraine de la France. Ces conséquences étaient connues de celles et de ceux qui ont voté la motion. Les 331 députés concernés doivent désormais s’en expliquer, au lieu de s’offusquer des effets d’une censure qu’ils ont célébrée. ! Pendant que nous prenons sur l’agenda parlementaire pour un tel texte, le temps court, avec son lot de défis et de difficultés. Pour l’heure, mes chers collègues, à nous d’adopter au plus vite ce projet de loi spéciale, que notre groupe votera évidemment, et de nous tenir prêts

devoir voter ce texte par nécessité, parce que la France n’aura pas réussi à se doter d’un budget au 1 janvier, constitue l’épilogue cruel d’un chantage à la motion de censure dont l’issue ne faisait guère de doutes : « La bourse ou la vie ! », en somme. J’y vois surtout un échec collectif, dont je prends ma part. Nous pouvons nous interroger sur la responsabilité des uns et des autres ; celle des parlementaires, celle du Gouvernement, celle du Président de la République et celle des institutions.

Le tragique dans cette histoire est que cet échec pourrait n’être que la première étape de la chute d’un régime vieillissant, affaibli et cerné par les populismes. Le piège se referme lentement sous nos yeux. Le régime s’enfonce tout seul dans une nasse bien tendue, affaibli par l’avachissement de ses institutions et par l’usage qui en est fait. affaibli aussi parce que la comptabilité et la gestion des risques ont supplanté l’humain et les idéaux politiques, à mesure que la bureaucratie a pris le pas sur les élus. Partout dans le monde, la victoire des populistes se fait contre les. Cette situation doit nous interpeller. Évidemment, le groupe RDSE votera en faveur de cette loi spéciale, afin de permettre un fonctionnement minimal de l’État. Mais nous appelons de nos vœux la convocation en urgence d’une conférence budgétaire, pour qu’une majorité arithmétique de parlementaires volontaires se constitue et fasse face à quelques points d’achoppement essentiels, avant de reprendre l’examen du budget 2025. Cette conférence doit être la plus large possible. Le dialogue doit réunir les démocrates de toutes les familles politiques, qui accepteront de considérer en priorité l’intérêt des Français. En effet, c’est bien d’eux qu’il s’agit Les dernières prévisions de l’Insee, il y a deux jours, sont alarmantes. En 2025, la croissance sera très affaiblie, si la commande publique ralentit. Les exportations seront fortement concurrencées par la production chinoise. Le logement et l’immobilier s’enfoncent déjà dans la crise. Les agriculteurs, comme vous le savez, sont aux abois. Chacun comprend qu’il sera impossible de construire un budget satisfaisant pour tout le monde, mais la gravité de la situation exige que nous trouvions un accord minimaliste, le moins mauvais possible. Concéder une victoire au compromis, en pareil cas, n’a rien de déshonorant.

Soyons lucides, mes chers collègues : notre vie politique continuera d’être traversée par des combats qui s’amplifieront, par des désaccords très profonds et par le retour des idéologies, qui viendront percuter les défis actuels : le mur de la dette, le changement climatique, la mondialisation et le financement du système de protection sociale. Serons nous capables de faire surgir de la mêlée des solutions démocratiques,

Premièrement, nous avons besoin de continuité, mais surtout de stabilité et de visibilité en matière de finances publiques. Ce projet de loi spéciale, dont nous nous félicitons, ne nous offre qu’une continuité partielle.

Mais demeurent de multiples incertitudes. L’effet de la censure sur le PLFSS et sur le PLF nous conduit à ajouter une zone de risque à une situation financière et politique déjà très critique. Autant dire qu’il y a urgence à reprendre

le seul remboursement des intérêts menace le pays d’étouffement et obère sa capacité d’action. L’assainissement de nos finances publiques est bien sûr un impératif. Ce projet de loi ne règle rien de ce point de vue. Troisièmement, nous devons retrouver une cohérence économique et financière. Là encore, cela passe par un par un projet de loi de finances. Il faut nous adapter à un contexte qui a changé, admettre que les 5 % de déficit seront difficilement atteignables, mais rester en cohérence avec nos engagements européens. L’incertitude est notre ennemie : elle pèse sur ce qui nous reste de croissance. Il nous faut parvenir à un ajustement budgétaire qui devra être dosé. Un ajustement budgétaire bien réalisé réduit l’incertitude et favorise la croissance ; un ajustement budgétaire mal dosé affecte fortement cette La baisse des taux et la maîtrise de l’inflation sont évidemment des éléments positifs, mais ils ne compenseront pas nos difficultés. Quatrièmement, et enfin, nous devons faire un effort collectif de responsabilité. Le projet de loi de finances ne correspondra pas à l’entièreté des positions de chacun, mais nous devons trouver les termes d’un compromis. L’économie, en effet, n’attend pas : les déficits continuent de se creuser. Le monde ne s’arrête pas : il évolue de plus en plus vite. La paralysie politique n’est pas compréhensible à l’heure où les défis sont nombreux.

Nous débattons aujourd’hui sous la pression d’une crise profonde et exceptionnelle. Et ce sont deux ministres démissionnaires qui présentent un texte qui fait office de budget pour la France ! Où est le Premier ministre ? La crise institutionnelle découle d’une crise démocratique qui couve depuis des années et qui explose aujourd’hui. Cette crise a un responsable : le président Emmanuel Macron.

Après cinquante jours de gouvernement démissionnaire, il confie le pouvoir à un Premier ministre issu d’un parti plafonnant à 5 % aux élections législatives, rendant inéluctable, par cette offense au suffrage universel, la censure de Michel Barnier. Le budget Le budget présenté pour 2025 était un budget de continuation du macronisme, aménagé un peu en bien, mais surtout en mal. La censure par l’Assemblée nationale, seule réponse possible au 49.3, était un acte politique fort et nécessaire, et notre force politique l’assume. Ce projet de loi spéciale aurait pu être présenté dans le cadre d’une nouvelle séquence où le Président de la République aurait enfin tenu compte du dernier en nommant une ou un Premier ministre issu de la force arrivée en tête aux élections législatives, pour ensuite, au Parlement, avancer texte par texte. Malheureusement, Emmanuel Macron, conseillé par ses mentors de la finance, s’est enfermé dans ses certitudes ultralibérales. Il a choisi de continuer vaille que vaille, sans rien changer, en foulant aux pieds les bulletins de vote, consacrant le coup de force démocratique enclenché le 9 juin dernier. Il faut changer de logiciel, il faut ouvrir en grand les vannes de la démocratie, construire une loi de finances pour 2025, avec et pour les citoyennes et les citoyens la mettre en débat partout, dans les métropoles comme dans les bourgs et les villages, sur les lieux de travail, avec les organisations professionnelles et avec les 250 000 salariés dont les emplois sont menacés.

Ces mensonges ont sali le débat politique : oui, ils ont sali le débat politique ! Et l’heure de la vérité a sonné. Cette loi spéciale vise à assurer la continuité de l’État et des services publics, et c’est tout. Pour la clarté de nos débats, je redis notre profond rejet du précédent projet de loi de finances.

Voilà le résultat du flou de l’article 45 de la Lolf ! Il n’est pas acceptable que les parlementaires, avant de voter la loi spéciale, ne connaissent ni la nature ni le montant global des crédits qui seront ouverts. Il est impératif de ne pas ajouter à l’incertitude politique une incertitude budgétaire. Il est frappant, à l’heure où chacun vante le parlementarisme, que députés et sénateurs se voient privés de leur droit d’amendement.

Le peuple français a raison de continuer à espérer vivre mieux, malgré les mauvais coups du président Macron et de la finance. Oui, le groupe communiste continuera à demander l’abrogation de la réforme des retraites et la revalorisation des salaires ! Comme l’écrivait si bien le poète Pablo Neruda : « Ils pourront couper toutes les fleurs,

Alors que, selon le calendrier initial, nous aurions déjà bouclé le projet de loi de finances 2025, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner un texte spécial, mais vital en ces temps troublés, le projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi Ce texte a vocation non pas à réorienter les grandes lignes de notre politique budgétaire, mais à garantir le fonctionnement de l’État dans une période d’incertitude. Il permet la collecte de l’impôt, le paiement des fonctionnaires et des pensions de retraite et la continuité des services publics, sur la base des services votés pour 2024. Un tel

Cette loi spéciale, nécessaire par sa nature, n’en demeure pas moins le symptôme aigu d’une crise politique et budgétaire majeure. Ne cherchons pas trop loin les responsables : la situation budgétaire catastrophique de la France en 2025 est la conséquence de sept ans de votre politique économique, messieurs les ministres

ministre de l’économie, Bruno Le Maire, ont appliqué sans relâche, jusqu’à l’absurde, une politique de l’offre, multipliant les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux ménages les plus aisés, sans jamais exiger de contrepartie, quelles que soient les crises que traversait le pays. le résultat de ces milliards d’euros pour quelques uns et de ces cadeaux fiscaux financés par la dette : 9 millions de pauvres, des plans sociaux qui se multiplient, nos collectivités qui se demandent comment boucler leur budget, un pays désarmé face aux catastrophes climatiques et le chaos qui envahit nos services publics sous financés. Cette crise budgétaire s’est transformée en crise politique, résultat d’un aveuglement politique qui vire au déni. La censure du Premier ministre Barnier est le dernier épisode en date de ce qui ressemble à une véritable débâcle institutionnelle due à un entêtement à poursuivre une politique dont la légitimité n’a plus de base démocratique. En nommant François Bayrou Premier ministre maire, le Président de la République s’enfonce dans le déni. déni. Nous le répétons, les mêmes causes produiront les mêmes effets : les mêmes ronds de jambe à Marine Le Pen et le même mépris pour la coalition de gauche arrivée en tête aux législatives aboutiront à la même chute de M. Bayrou.

le Gouvernement, dans son mépris habituel, a préféré imposer de secondes délibérations pour balayer les nouvelles recettes que nous avions inscrites dans le projet de loi. Osons donc un conseil : dans l’intérêt du pays, le mépris du travail parlementaire doit quitter Bercy dans les valises des ministres démissionnaires. Cette loi spéciale, si elle est nécessaire pour éviter le chaos, n’est qu’un palliatif. pays a besoin d’un véritable budget qui soit à la hauteur des défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels nous faisons face. Nous, écologistes, appelons de nos vœux budget fait de priorités claires et de réels investissements dans la transition écologique, qui organise la solidarité et qui redonne des moyens à nos services publics, le tout financé par la justice fiscale. Mes chers collègues,

des 5 % de déficit à la fin de 2025, un objectif que Michel Barnier et son gouvernement, dont je veux saluer l’action, s’étaient engagés à tenir. L’urgence budgétaire L’urgence budgétaire demeure donc et va même s’amplifiant, dans une déliquescence politique qui semble ne jamais s’arrêter. Je me réjouis pourtant que, au désordre de nos comptes et à l’incertitude politique du moment, on n’ajoute pas une aventure juridique. soit un État de droit, disposant encore d’institutions fortes et d’un système administratif efficace, voilà sans doute le dernier signe de la crédibilité et de la stabilité de notre pays ; ne le galvaudons pas

Notre économie est en panne. Les nouvelles prévisions de croissance sont bien inférieures au 1,1 % escompté pour 2025. Les défaillances d’entreprises se multiplient. Patronat et syndicats s’unissent pour alerter sur les risques d’une crise économique aux conséquences sociales dramatiques. Par delà cette loi spéciale, qui agit comme un respirateur artificiel, nécessaire mais limité, il faut traiter l’urgence budgétaire sur le fond.

ce n’est pas d’un projet de loi portant diverses mesures économiques et financières et mettant la question budgétaire sous le tapis – cela, c’est ce que demandent ceux qui ont empêché le PLF d’aboutir.

Je ne veux pas agiter le chiffon rouge du chaos : la peur n’est jamais bonne conseillère et elle est souvent contraire au bon sens, des expériences récentes l’ont encore montré. Je crois davantage à la pédagogie et je veux faire confiance à l’intelligence de chacun, ainsi qu’à notre intelligence collective. je sais aussi que, comme l’écrivait Tocqueville, « ce qu’il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c’est ce qui se passe sous nos yeux ». Formons le vœu que nous sachions voir clair et loin dès le début de l’année 2025,

Certes, en 1979, il y a quarante cinq ans, un texte similaire avait été soumis au Parlement, mais le contexte était très différent : il s’agissait uniquement d’un problème de procédure, qui avait conduit le Conseil constitutionnel à annuler la loi de finances, laquelle avait pu être promulguée dès le dès le 18 janvier suivant. La situation n’est malheureusement pas de même nature aujourd’hui, puisque nous terminerons l’année sans loi de financement de la sécurité sociale, sans loi de finances, sans réelle visibilité sur le calendrier dans lequel ces textes pourront être adoptés, et sans gouvernement. Cette loi spéciale est donc indispensable pour éviter la paralysie totale de l’État et permettre son bon fonctionnement minimal. Pour autant, elle ne réglera pas tout, tant s’en faut. Malgré son adoption, de nombreuses difficultés demeureront jusqu’à la promulgation de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale, qui n’interviendront probablement pas avant plusieurs mois. Je voudrais, à cet égard, souligner l’irresponsabilité de ceux qui ont voté cette motion de censure, qui n’a que des effets négatifs pour la France et les Français. Elle aura des conséquences sur 18 millions de Français, qui verront leur impôt sur le revenu augmenter ou qui deviendront assujettis à cet impôt. Elle privera, pour plusieurs mois, les agriculteurs de mesures financières attendues, les forces de l’ordre de moyens supplémentaires, la Nouvelle Calédonie des crédits dont elle a besoin pour se reconstruire. Je pourrais également évoquer les conséquences de cette motion sur le chèque restaurant, le prêt à taux zéro et la prise en charge des frais de transport Je pourrais aussi, et surtout, évoquer les conséquences économiques et financières de cette censure. La dégradation de la note de la France par l’agence Moody’s en est le premier signe et vient renforcer les inquiétudes des investisseurs et des consommateurs. Quant aux collectivités locales, elles vont – pour la première fois – commencer l’année sans la moindre visibilité sur les concours dont elles bénéficieront pour mettre en place leur budget. Il ne sera pas facile de l’établir dans ces conditions

ci devra, de mon point de vue, proposer plus d’économies que le projet de loi de finances initial, qui comptait trop de hausses de fiscalité et pas assez d’économies. Vous y allez fort ! Je comprends que les délais contraints qui ont été imposés au gouvernement de Michel Barnier et qui s’imposeront à celui de Français Bayrou rendent la tâche particulièrement difficile. C’est pourquoi j’en appelle au Gouvernement pour que, dès maintenant, il s’attelle, en vue du budget pour 2026, à une revue générale des dépenses publiques, qu’il interroge ligne par ligne, euro par euro, l’utilité de chaque dépense, comme nous savons le faire dans nos collectivités. De toute évidence, il existe des économies potentielles importantes parmi les nombreuses agences de l’État qui se sont multipliées au fil des ans ou dans la gestion du parc immobilier de l’État, qui doit être rationalisée. Le pilotage des ressources humaines doit également être optimisé

que nous n’avons pas souhaitée. La situation dans laquelle nous avons été entraînés nous oblige à faire cette sorte de faux témoignage

Sans entrer dans les détails, et pour n’évoquer que l’article 3, je vous invite, mes chers collègues, à mesurer avec moi les effets néfastes

Pis encore, ils ont envoyé aux négociations complexes et difficiles du Mercosur un pays affaibli, avec un gouvernement démissionnaire. Ceux qui prétendent « avoir le monopole du cœur

d’un certain nombre de dispositifs urgents en leur faveur ou en faveur des structures médico sociales qui les accueillent ! En matière de santé, leur comportement a retardé la lutte contre les déserts médicaux, la mise en place de mesures de prévention sanitaire, la lutte contre la fraude sociale et l’amélioration de la pertinence de l’offre Mes chers collègues, cette loi spéciale dans le contexte actuel est une étape obligatoire. Mais cette solution technique et juridique que nous serons contraints d’adopter ne doit pas valider la notion de, qui conduit sans nul doute à aggraver le déficit. le déficit. La maison brûle, ne restons pas aveugles ! Pour ma part, je reste confiant en notre capacité à réagir et à ne pas occulter les problèmes de fond qu’il est urgent d’aborder

L’État français doit déployer tous les moyens possibles pour leur venir en aide et permettre leur deuil : tout est à reconstruire. L’objet de mon intervention dans le cadre de l’examen de cette loi spéciale est la situation de la Kanaky Nouvelle Calédonie. si la loi de fin de gestion a ouvert des crédits supplémentaires pour le pays, le projet de loi de finances est quant à lui en suspens. Le débat budgétaire sur les crédits de la mission « Outre mer » aurait été pour moi l’occasion de m’opposer à la logique de prêts envisagée pour la Nouvelle Calédonie.

dans un contexte d’endettement de plus de 340 %. Avec de tels prêts, l’endettement de la Kanaky Nouvelle Calédonie aurait alors Quelles perspectives de développement reste t il à un territoire endetté à un tel niveau ? Il y a urgence à reprendre les débats budgétaires, pour apporter des réponses à la hauteur des besoins pour le début de l’année 2025.

! L’audiovisuel public est financé désormais un compte de concours financiers, abondé pour 2025 par un amendement au Sénat, donc en cours de discussion dans le cadre du projet de budget abandonné. Il aurait pu faire l’objet d’un prélèvement sur recettes exceptionnel pour assurer la continuité du service public sans contrevenir à la loi organique du 13 décembre 2024 portant réforme du financement de l’audiovisuel public. De même,

avait été déclarée recevable en 1979, lors du seul précédent rencontré à ce jour en matière de discussion d’un projet de loi spéciale.

Monsieur le président, messieurs les ministres démissionnaires, ce texte est issu d’un contexte politique suscité par l’irresponsabilité : celle du Président de la République, qui n’entend pas nos territoires ; celle du Premier ministre Barnier,

ici au Sénat comme lors de la commission mixte paritaire, des propositions responsables pour réduire le déficit de notre sécurité sociale et pour garantir l’avenir de notre système de protection sociale. Ce rejet de notre main tendue au Gouvernement a conduit au rejet du PLFSS et à la censure. Le sujet des recettes n’est pas tabou, et nous devons reconsidérer les exonérations de cotisations sociales lorsqu’elles sont inefficaces pour l’emploi et pour la compétitivité des entreprises. Nous devons assurer plus d’équité par la contribution des plus aisés à nos dépenses de santé, des recettes indispensables pour assurer la protection de nos concitoyens, de la crèche à l’Ehpad, en passant par l’hôpital. Ce projet de loi spéciale prévoit la possibilité pour l’Acoss d’emprunter, donc de financer les caisses de sécurité sociale autant que nécessaire. qu’il soit indispensable, ce texte ne répond pas à l’exigence qui s’impose à nous de répondre aux agriculteurs attendant une revalorisation de leur retraite, aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et aux professionnels de santé. spéciale n’est pas une loi de financement de la sécurité sociale. Elle risque même d’aggraver les déficits. Puisqu’elle répond toutefois à l’urgence et à l’instabilité dans laquelle nous a plongés le Premier ministre Barnier, nous la voterons. Il n’empêche que la situation nous oblige, en responsabilité, à reprendre le travail engagé, pour que chacun contribue équitablement à ce budget et pour que chacun puisse être assuré d’une prise en charge de qualité,… C’est fini ! … ce qui n’est plus le cas dans notre pays, qui est confronté à des difficultés d’accès aux soins et à la détresse de nos hôpitaux. Nous sommes prêts à y travailler et à réitérer nos propositions au futur gouvernement Bayrou, afin de répondre aux préoccupations exprimées par les Françaises et les Français dans les urnes.

Si le Premier ministre avait été là, nous lui aurions réitéré notre souhait qu’il y ait bien un nouveau budget et que l’on ne reprenne pas les travaux parlementaires comme si rien ne s’était passé. Nous allons donc voter favorablement, mais il faut revoir la copie. La

avec les mêmes conséquences ? Ou allez vous enfin comprendre et infléchir votre politique avec un peu plus de justice fiscale, un peu plus de justice sociale, un peu plus d’égalité, un peu plus de partage dans notre pays ? Personne

Le scrutin est ouvert.

J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi du 23 juillet 2010 la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable, par vingt voix pour et neuf contre, à la nomination de Pierre Monzani à la présidence de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Par ailleurs, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a émis un avis défavorable, avec douze voix pour et dix sept voix, contre à la nomination de M. Martin Ajdari à la présidence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.